La séance est reprise en application du 5ème alinéa de l'article 13 de la Constitution. Ainsi que de la loi organique. Et de la loi ordinaire, numéro 2018 138 du 23 juillet 2010 prises pour son application. La commission des finances a émis lors de sa réunion de ce jour un avis favorable. 19 fois pour aucune voix contre à la nomination de monsieur Éric Lombard aux fonctions de directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. L'ordre du jour appelle le débat sur les conclusions du rapport, faire de la RS. Une ambition et un atout pour chaque entreprise demande de la délégation aux entreprises. Je vous rappelle que dans ce débat, le gouvernement aura la faculté s'il le juge nécessaire. De prendre la parole immédiatement après chaque orateur pour une durée de deux minutes. L'orateur disposera alors à son tour du droit de répartis pour une minute s'il le souhaite. Madame la Ministre, vous pourrez donc si vous le souhaitez répondre après chaque orateur, une fois que celui-ci aura retrouvé une place dans l'hémicycle. La parole et tout d'abord aux orateurs de la délégation aux entreprises qui a demandé ce débat. Madame Martine Berthet au nom de la délégation aux entreprises. Ensuite ce sera monsieur Jacques Le Nay au nom de la délégation aux entreprises puis Madame Florence. Ce compta toujours au nom de la délégation. Madame Berthe et vous avez la parole. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. La responsabilité sociétale des entreprises s'inscrit dans une nouvelle grammaire de l'économie. Elle affecte profondément les modalités de production et de commercialisation et constitue un enjeu de pouvoir au sein des grandes entreprises cotées. Ces dernières sont les principales cibles de la législation tant européenne que nationale et de la soft law international des normes et labels, dont le rapport de la délégation aux entreprises de juin 2020 avait souligné le caractère foisonnant. Nous avions alors proposer d'harmoniser le Champ d'application des obligations de publication de données extra-financière d'éviter les informations redondantes et de se focaliser sur celles qui sont significatives. Le choc de complexité en matière de RSE que nous avons relevés dans le 2ème rapport d'octobre 2022, adopté à l'unanimité est un défi pour les grandes entreprises, comme l'a souligné l'autorité des marchés financiers en décembre 2021. Que dire alors pour les PME, car elles sont aussi concernées directement ou indirectement lorsqu'elles appartiennent à des chaînes de valeur, ce qui est souvent le cas. Personne n'a chiffré le coût humain et financier que représente l'obligation pour elle de fournir un volume d'indicateurs toujours plus important toujours plus complexes toujours plus redondants. Le projet de standards de les fringues groupe consultatif européen sur l'information financière comptait 130 items, c'est trop. D'autant que ces indicateurs seront complétées par des informations spécifiques à chaque branche les normes européennes ou nationales doivent s'appliquer très progressivement aux PME et ce rythme doit prendre en considération l'environnement économique très dégradé actuellement. N'ajoutons pas à l'inflation monétaire une inflation réglementaire ce mille-feuille doit être simplifié, sinon il sera indigeste. Le rapport de la délégation aux entreprises proposent un principe de proportionnalité, fonction de la taille et des moyens de l'entreprise. Sans oublier le respect de la confidentialité de sa stratégie, principe qui devrait se décliner par une approche sectorielle différencie. Enfin et surtout, nos entreprises doivent pouvoir se battre à armes égales et veiller à ce que les entreprises non européennes soient soumises à des exigences équivalente en matière de publication d'informations extra-financière, c'est une condition de la durabilité de la compétitivité de nos PME. Monsieur le nez, vous avez la parole. madame la présidente. Madame la ministre de l'énorme sont un enjeu essentiel de la souveraineté pour les entreprises. La norme c'est la notation et la notation, c'est l'accès au crédit, voire au marché. Cette loi s'applique particulièrement la RSE et à la publication d'informations que presque toutes les entreprises devront prochainement produire pour évaluer leurs performances guidées les choix de gestion de leurs dirigeants et orienter les investissements. Au début des années 2000, l'Europe avait perdu la bataille des normes comptables et les standards américains se sont imposés une nouvelle défaite ne peut être subi. D'autant que les normes et les entreprises européennes sont en avance dans ce domaine, l'Europe étant le continent d'un capitalisme plus responsable dans le rapport de la délégation aux entreprises adoptée en octobre dernier, nous avons pointé 3 défis. Le 1er celui d'un standard unique des critères ESG. Car un double standard mondial créerait une complexité inutile à cet effet, le dialogue entre les 3 entités que sont le groupe consultatif européen sur l'information financière, le Bureau international des normes comptables et le gendarme américain de la bourse doit déboucher sur un pacte mondial avec des normes dit des recommandations communes. Le 2ème défi est celui du contenu de l'information permettant d'évaluer la performance d'une entreprise. Son évaluation ne peut plus se baser uniquement sur ses performances économiques et financières, mais doit obtenir compte de son comportement vis-à-vis de l'environnement. Du respect des valeurs sociales et de l'éthique. De son engagement sociétal et de son gouvernement d'entreprise, il y a donc pas d'un côté l'information financière et de l'autre l'extra-financière cela suppose l'abandon de la conception Friedman viennent de l'entreprise qui ne peut se réduire à la seule création d'un d'un profit. Il y a encore des esprits à faire évoluer sur ce terrain, notamment aux États-Unis. Enfin 3ème défi, celui de la reconquête de l'autonomie et de la souveraineté en matière de notation et de publication des données des entreprises. Les agences de notation européenne sont toutes passées sous contrôle américain. Leur méthodologie respectifs diffère la nouvelle directive si SRD. Permet une harmonisation européenne. Bienvenue. Comme le recommandait l'Autorité française des marchés financiers en mars 2021. L'Autorité européenne des marchés financiers doit devenir le point d'accès européen unique pour les données financières et extra-financière des sociétés cotées. Où en est cette proposition. Merci monsieur le nez. La parole est à madame Blétry. Ce constat. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues la ARS doit être un atout pour chaque entreprise car elle porte en elle l'exigence de la transition climatique. La réduction des gaz à effet de serre étant l'un des indicateurs de performance environnementale, sociale et de gouvernance dites ESG à cet effet le rapport Perrier de mars 2022, qui souhaite faire de la place de Paris, une référence pour la transition climatique propose comme la délégation l'avait évoqué dès juin 2000 bas d'instaurer une comptabilité carbone quelles suites ont été données à cette proposition. Ainsi que nous l'avions recommandé dans le rapport de la délégation aux entreprises adoptée en octobre dernier. Le MEDEF préconise dans sa nouvelle version de son code de gouvernance que la RSE soient placés au coeur des missions. Du conseil d'administration des entreprises cotées deviennent un élément important de la rémunération de leurs dirigeants mais il recommande que les orientations stratégiques pluriannuels ne soit présenté que tous les trois ans et que la formation des administrateurs sur les enjeux RSE soit une possibilité. Seulement il faut être plus ambitieux, notamment pour la formation des salariés, administrateurs qui devrait être entre un droit voire une obligation pour être durable, la démarche RSE des entreprises doit être crédible. Or la publication d'une enquête de médias européens fin novembre a confirmé les craintes. À la notion des craintes relatives à la notion de finance durable que nous avions évoqué dans notre rapport déjà le rapport de l'Inspection générale des finances sous le Label public. ISR investissement social et responsable, appelait à la réforme. La présidente du comité du Label ISR s'y attelle depuis mars 2021, ces orientations sont attendus. Pouvez-vous nous en dire plus. Cette réforme semble d'autant plus urgente que l'enquête journalistique a souligné que la moitié des fonds dits durables, y compris les fonds super verts investissait encore dans des énergies fossiles en contradiction flagrante avec la réglementation européenne. Pourtant, en mars 2020, le ministre de l'Économie, indiquait qu'il fallait l'assurance que la finance verte ne soit pas du greenwashing cela relève nom cela Cela révèle non seulement l'hétérogénéité des notations EG mais interroge également sur la crédibilité des engagements climatiques de certaines entreprises, remet en question le modèle de l'audit des entreprises financières ou non. Les professionnels du chiffre capable de décrypter, de vérifier la comptabilité financière des entreprises seront-ils désormais capable d'évaluer la sincérité d'engagements sociaux, environnementaux, sans formation spécifique, quel rôle doit être dévolu aux experts comptables interlocuteur privilégié des PME. Par ailleurs, un immense chantier de formation doit s'ouvrir comme le propose le rapport pour rendre obligatoire pour tout ce qu'il se destine au monde de l'entreprise. La formation aux enjeux de l'ARS. Vous mais nous vous remercions. Madame la Ministre. Espérons que ce sujet sera portée au-delà de ce débat parce que c'est un sujet important pour nos entreprises elles attendaient pour notre économie. Je vous remercie. Si cher collègue dans la suite du débat. La parole est à monsieur Thomas dessus. dessus. Pardonnez-moi, monsieur le sénateur, je serais rapide le chronomètre en attestant. Bonsoir à toutes et à toutes. Bonsoir madame la vice-présidente. L'occasion de vous retrouver et je prends sur mes deux minutes pour vous souhaiter très très vite une très belle emmener avec la santé, la joie puisqu'on y a droit. Malgré les difficultés et j'enchaîne très vite. Mesdames, messieurs les sénateurs pour vous remercier vous remercier malgré l'horaire tardif malgré les différentes urgence majeure qui nous occupe tous. Je veux vous dire à quel point je suis reconnaissante d'avoir pris le temps de produire un rapport aussi intéressant approfondie que celui qui a commis la délégation sénatoriale aux entreprises et surtout d'avoir pris le temps de tenir ce débat ce soir sur un sujet absolument essentiel pour la compétitivité de nos entreprises, pour avoir été pendant plus de deux ans secrétaire d'État à l'économie responsable. Je sais bien ce qu'on dit de la responsabilité sociale de nos entreprises, c'est très très bien c'est très très important, mais ça n'est pas vraiment l'urgence tout le monde et donc d'accord. En un mot qu'il faut faire quelque chose, mais en réalité, ça n'est jamais vraiment le bon moment votre présence ce soir votre mobilisation au sein de la délégation démontre que nous devons affirmer le contraire. Vous avez tous les trois en introduction abordé de nombreux sujets qui demanderait et c'est frustrant. Un peu plus de deux minutes des deux minutes dont je dispose et je vais vous dire que je ne pourrais pas toujours apporter des réponses exhaustives. Dans ces deux minutes, compte tenu de, de l'exode. Invité des sujets de leur profondeur mais que je prends l'engagement devant vous devant la délégation mais devant chacun des sénateurs et sénatrices de prendre le temps de vous répondre plus en profondeur si je ne peux pas tout détailler dans le temps qui m'est imparti. Je veux avant tout aussi profité de ce propos liminaire pour vous partagez l'état d'esprit qui est le mien. La France et vous l'avez dit, la France et l'Europe avance à grands pas sur ces sujets de RSE. La France est en avance. Il nous faut préserver notre avance. Il nous faut aussi accompagner toutes nos entreprises. Les grandes, les entreprises de taille intermédiaire sont directement concernés par le Champ de la directive CSR dès que vous avez mentionnées nos PME le seront, vous l'avez très bien dit directement ou indirectement, la question c'est comment et comment proportionnellement on accompagne, chacune d'entre elles. J'ai à coeur de vous répondre aussi exhaustivement que possible. Je vous remercie. Merci madame la ministre et donc la parole est à monsieur Thomas Dossus pour le groupe écologiste solidarité et territoires. Oui, très rapidement. Merci madame la ministre. Ce sur quoi nous souhaitons vous alerter également c'est sur la sur-transposition qu'il risque d'y avoir de la directive européenne donc une transposition qui se fera vraisemblablement sous forme d'ordonnances et nous souhaiterions être être associés à ce travail. De façon à ne pas être dans la surtransposition. C'est important pour les entreprises. Je vous remercie. Merci madame Berthe et monsieur dessus. Merci madame la présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues. Donc là et Racer et ce peu stabilité sociétale et environnementale des entreprises c'est basiquement la prise en compte des enjeux de développement durable environnementaux, sociaux et et de gouvernance par les entreprises parfois caricaturé en saupoudrage de bonne conscience entre entrepreneuriale ARS et le dépassement de la logique purement comptable ou financière et la prise en compte des logiques responsable des entreprises une armée une amélioration cette notion a été rendue nécessaire, voire indispensable, ces dernières années, car la nature même des entreprises n'est pas fondamentalement sensible aux 3 piliers du développement durable, l'ARS est un mouvement complémentaire complémentaire au mouvement social et écologique, un élan, cette fois-ci destiné principalement aux consommateurs, aux investisseurs et au monde associatif, l'amélioration des normes RSE doit rendre les entreprises vertueuses, les plus vertueuses, les plus compétitives. La société a des attentes de plus en plus forte vis-à-vis des entreprises, elle attend de celle-ci que leur impact environnemental soit le plus réduit possible voire même soyons ambitieux que celui-ci soit positif que l'entreprise traite non seulement bien ses employés, mais aussi qu'elle soit vigilante sur son impact global la rationalité économique ne doit plus être les l'ennemi du vivant. Si la RSA a été à ses débuts. Un mouvement volontaire de la part des entreprises. Nous sommes aujourd'hui dans une phase plus contraignantes et heureusement plus exigeante, plus contraignante, notamment par l'édification de normes et de référentiel commun à ce titre et le rapport dont nous examinons les conclusions aujourd'hui le souligne très bien l'Europe est un continent en pointe sur ces questions. C'est ainsi l'Union européenne qui était à l'origine en 2013 de la déclaration de performance extra-financière pour les grandes entreprises complété par la directive N F R D en 2018 faisant partie de la taxonomie verte européenne extra- financière doit inclure des informations. Sur l'entreprise relatives aux questions environnementales aux questions sociales et de personnel, de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption, c'est également l'Europe. Qui décide d'assujettir les grandes entreprises au devoir de vigilance. Et qui c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui a mis en avant le concept de double matérialité. Dans la directive c'est SRD ce concept de double matérialité est assez avancé, puisqu'il prévoit que les entreprises devront non seulement à examiner les conséquences de la dégradation des conditions sociales et environnementales sur leurs activités mais aussi mesurer la manière dont l'activité de l'entreprise influe sur ces mêmes conditions dans une double relation de cause à effet. Ces directives s'accompagne principalement d'obligations nouvelles en terme de reporting. C'est ce qui inquiète particulièrement les entreprises et c'est principalement ce à quoi répond le rapport que nous examinons aujourd'hui dans les proportions dans les propositions avancées par nos rapporteurs nous trouvons tout d'abord la nécessaire proportionnalité des exigences en matière de RSE, qui doivent être imposées selon la taille de l'entreprise, on ne demande pas la même chose à une PME ou à une multinationale et cet objectif s'entend parfaitement. Vient ensuite un souhait de renforcer. De renforcement du rôle de l'Autorité européenne des marchés financiers, un effort d'harmonisation des normes une montée en puissance de la formation ou encore l'introduction d'une notion d'offres écologiquement la plus la plus avantageuse dans le code des marchés publics. Notre groupe écologiste salut naturellement ces propositions qui vont dans le bon sens et propose des ajustements bienvenue à la montée en puissance de l'ARS. Si le reporting et la transparence sont des ET nécessaire de régulation et d'information des. Des consommateurs est parti. Prenantes en tant qu'écologistes, nous sommes convaincus que la solution réside aussi et surtout dans le changement profond de nos modes de production, de consommation et de gouvernance intégrer des logiques non financières dans la marge entreprise devient une évidence. En revanche. L'économie dans la limite planétaire ne l'ai pas encore communiqué comme le fait Total par exemple sur des objets qui sont des efforts de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, de moins 40% d'ici 2030, tout en continuant d'ouvrir des nouvelles exploitations et de rechercher de nouveaux gisements d'énergies fossiles et d'une hypocrisie rare qui nous conduit tous et toutes vers la catastrophe. Ce n'est pas la ARS qui ne sortira qui nous en sortira mais la contrainte publique le changement doit être plus profond, plus radicale, plus contraignant aussi et la RSE ne pourra pas ne pourra pas parvenir seul à changer les règles. Et ne peut suffire comme outil de régulation de l'impact du monde économique sur nos vies et notre avenir. Je vous remercie. Si cher collègue, madame la ministre. Merci madame la présidente. Déjà j'ai à coeur. Monsieur le. Le sénateur de. Remettre un peu en en perspective. L'ensemble des coalitions internationales sur laquelle la France a été plutôt moteur pardonner. Les multiples abréviations. Que ce soit la TNF dès la Task force sur le Finding sur le disque logeurs pardonnez l'anglais mais c'est aussi en anglais, que ce soit aussi. L'ADN FD à laquelle j'imagine que vous êtes. Particulièrement sensible, la task force nature donc à destination de notre biodiversité avec un travail de titan qui est en train d'être menée. Et et c'est un travail et d'ailleurs passionnant. À l'endroit des des ressources naturelles de notre planète et de nos espèces et la façon dont l'activité économique impacte notre nature et la biodiversité. Il a donc énormément de coalition. Mondiale qui sont aujourd'hui pour partie impulser si ce n'est nourri alimenté beaucoup par la France qui est moteur en Europe pour y avoir siégé y avoir contribué pendant 2 ans au moins au côté du président de la République. Je pense qu'il nous faut aussi être vigilant sur ces coalitions parce que c'est comme toujours trop de coalition si vous me pardonnez-nous perdent aussi un peu parfois et pour ne pas dire tu les coalitions. Je fais donc très attention depuis Bercy avec Bruno Lemaire. Est-ce qu'on empile pas des coalitions. Qui en réalité sont forts de déclarations d'intention, plutôt que d'actes ferme. Et je pense qu'il nous faut quand même avoir cette vigilance tous ensemble avec les parlementaires sur la proportionnalité. Que vous avez mentionnées. C'est pas la même histoire pour une grande entreprise, une entreprise de taille intermédiaire et une PME. C'est un défi d'y répondre en 22 secondes. Je veux juste vous dire. la la directive CSR des mais on aura l'occasion j'imagine d'en reparler s'applique au moment où on se parle uniquement aux entreprises de plus de 250 salariés dans le périmètre européen donc aux PME. Non cotées uniquement pour ce qui concerne les entreprises de taille PME donc j'aurai l'occasion d'en reparler, je suis acquise à la proportionnalité. Encore une fois c'est une déclaration. Maintenant il faut qu'on vérifie dans les actes et surtout dans les actes délégués qui vont nous arriver que cette proportionnalité est effective, je vous remercie. Merci, madame la Ministre. Pas de réplique merci messieurs dessus. La parole est à monsieur Jean-Baptiste Lemoyne pour le groupe RDPI. Bien, madame la présidente, monsieur le président de la la délégation. Mesdames les membres. Monsieur le rapporteur. Madame la Ministre naturellement. On se penche sur un sujet qui qui est très tendance. Mais je veux avant tout Thierry mon chapeau puisque le Sénat lui dans la constance. On est là sur un 2ème rapport et c'est important effectivement de suivre cette mise en neuf depuis les premiers travaux dans les années 50 60 sur ce thème depuis la prise de conscience à Rio. Dans les années 90. Eh bien force est de constater que il y a une ébullition une émulation collective. La France, c'est vrai. Prend toute sa part. Mais de façon, je pense positive pour être tout à fait objective. Avec l'article 116 de la loi NRE, on s'en souvient, les lois Grenelle 1 et 2 récemment. La loi pacte vous y avez contribué. Madame la ministre avec. Ce concept de société à mission par concept ce statut pour affirmer sa raison d'être. Mais c'est vrai il y a aussi le risque. D'un affichage parfois. Ça a été pointé par le rapport Rocher. D'où la nécessité au-delà des tendances de revenir à l'essence de ce qu'est la RSE. tout simplement que l'entreprise elle n'est pas une fin en soi mais qu'elle est un moyen. C'est simple, nous, citoyens, on a des droits et on a des devoirs, hé bien l'entreprise elle a accès à des libertés économiques. Mais là aussi des responsabilités économiques dont elle est redevable et c'est de bien, c'est bien de ça dont il s'agit. L'entreprise elle évolue dans Environnement. a un impact sur cet environnement positif comme négatif. C'est bien ce concept de double matérialité et on le voit bien sur le sujet des retraites, qui nous occupe aujourd'hui. Où en est-on sur l'emploi des seniors et ben on n'est pas là où on devrait être il y a une responsabilité sociale des entreprises, de ce point de vue-là c'est un peu dommage d'ailleurs de constater que, à chaque fois il faut y aller à coups de. De menace de quotas de sanctions pour parfois faire bouger les lignes. Je ferme la parenthèse. Mais d'où l'importance des perspectives tracées par le président de la République et des chantiers qui l'a annoncé. Je pense au chantier du partage de la valeur au chantier de la rémunération des dirigeants qui évoquait dans sa campagne conditionner aussi. Hé bien ce. Cette rémunération au respect des objectifs environnementaux et sociaux de l'entreprise peut-être sur ce point, de la Ministre pour nous éclairer sur la suite de la mise en oeuvre de cet engagement. Alors comment passer. Des principes généraux et généreux à une mise en oeuvre qui doit répudier tout angélisme parce qu'on est dans la compétition mondiale qu'on ne doit pas perdre de vue nos intérêts, les intérêts de nos entreprises, nos PME pour cela les accompagner. Alors effectivement recommandations de trois et quatre du, du rapport de la mission de la proportionnalité de la simplicité de la progressivité progressivité simplicité. On est avec la directive, c'est à cerner, entrée en vigueur. 2027 2028 pour les PME. Dénoncent spécifique sur lesquels travaillent les fringues pour les PME. Donc ça va dans le bon sens. D'ailleurs, de ce point de vue là je pense qu'il ne faut pas non plus. Retarder le moment dans lequel les PME. Se mettent dans cet état d'esprit parce que c'est une demande du consommateur, c'est une demande du citoyen, c'est une demande dans l'investisseur et donc c'est un service à leur rendre que de les aider à y aller. Et de ce point de vue là madame Bertrand, je pense que une petite occasion manquée ici au Sénat parce que. On aurait pu y aller avec l'article 8 du projet de loi Dadu. La la transposition de la directive, elle va permettre aussi des mesures de simplification. Il y a eu un rapport du Haut comité. Naturellement juridique de la place de Paris et puis la double matérialité elle t'affirmer par cette directive et on est là au coeur d'ailleurs des anges normatif au niveau mondial matérialité vision US versus double maille matérialité version européenne. Et c'est pourquoi ne soyons pas naïfs, on est dans ce monde de guerre économique. Les Américains, ils ne sont pas prévenu quand ils ont ils allaient faire leur une fashion réduction Act, hé bien nous de cette même. nous devons ne pas être naïf, il est heureux d'ailleurs que la directive c'est SRD permettent. Aux États d'autoriser des entreprises à omettre certaines informations quand il y a des intérêts commerciaux majeurs qui sont en jeu. Ça montre bien que, voilà on n'est pas des naïfs et puis ça veut dire prendre en compte aussi l'équité dans la concurrence. De ce point de vue là une des propositions du rapport, c'est d'assurer un traitement identique dans le reporting pour les entreprises non européennes recommandation numéro 5 j'y adhère. Nous devons y adhérer la directive d'ailleurs si cerner. De ce point de vue-là est un peu perfectible parce qu'elle elle ne le fait que pour les entreprises qui ont des filiales ou. Comment dire des succursales dans l'UE. pour la directive. Devoir de vigilance, on doit aller plus loin, je pense que la France d'ailleurs porte cette ambition et inclure toutes les entreprises étrangères qu'elles aient ou pas des filiales en en Europe parce que vous pouvez très bien faire des affaires, faire du chiffre d'affaires en Europe sans pour autant avoir des établissements qui sont sur le sol européen et puis encadrons aussi l'activité des agences de notation on l'on ça a été pointé par le rapport sont majoritairement sous contrôle américain. Nous pouvons introduire je crois une réglementation au niveau européen pour plus de transparence pour gérer aussi les problèmes de conflit d'intérêts. Pour superviser ces agences. De notation ESG par l'Autorité européenne des marchés financiers, donc en conclusion. Je dirais, garder notre avance effectivement la Ministre souligné. Cette avance française et européenne. Ne nous laissons pas faire d'ailleurs par ce qui, rappelez-vous, qui a voté contre la norme ISO 26.000 en 2010. Les États-Unis et Cuba sont retrouvés côte à côte hein c'est quand même une alliance assez improbable. Et donc notre spécialité européenne, nous devons la défendre gardant les valeurs qui sont eux au coeur de la RSE, celle de la dignité de l'homme du respect de notre environnement et d'ailleurs la préhistoire de la RSE. C'est assez comique quand vous regardez dans les textes, c'est à la fois prudent et le pape Léon XIII voilà l'auteur des contradictions du système économique et et celui de l'encyclique Rerum novarum tous les deux avaient à coeur le juste salaire et Simplement parce qu'ils avaient à coeur la dignité. Humaine et c'est bien ça, on a des enjeux qui sont supérieurs qui sont. Prioritaires, les ODD, c'est l'affaire de tous, 2030 c'est demain, alors c'est l'affaire de l'État. L'affaire des entreprises. Saluons le réseau France du Pacte mondial et les collectivités qui doivent embarquer naturellement parce que nous sommes tout simplement tous des pays en voie de développement durable. Donc on se retrousse les manches. Merci. Merci Monsieur Lemoine. Madame la ministre vous avez la parole. Merci madame la présidente. Si. Le ministre-Lemoine l'accepte. Je lui emprunterai cette expression, nous sommes tous des pays en voie de développement durable. Et même si la France n'est pas en reste n'est pas en retard, Pour se satisfaire des années et des. Progrès qu'on a pu faire tous ensemble. Que ce soit d'ailleurs au niveau des des parlementaires comme au niveau du gouvernement. Monsieur le député, le sénateur Lemoine a à relever. de nombreux points très intéressant dans la minute 30 qui mettent un parti j'aimerais répondre à votre sollicitations concernant. La corrélation qu'on pourrait mettre en oeuvre pour le dire simplement entre la rémunération des dirigeants et l'état de la performance extra- financière des entreprises qu'il dirige. Une recommandation que vous avez portée je crois que c'est celle qui est la numéro huit et vous dire. Que au-delà de cette corrélation entre la rémunération et l'état de la performance extra-financière de l'entreprise dirigée. Il y a les enjeux de formation des membres du conseil d'administration des comités de direction et j'irai même. Aussi jusqu'à intégrer évidemment les administrateurs salariés vous en avez dit un mot, madame la sénatrice, son introduction, la formation des administrateurs des mandataires sociaux et d'un levier essentiel c'est un débat que j'ai assez souvent moi aussi avec le MEDEF. Et je pense que vous le savez, mais je pense qu'il nous faut être vigilant, tous ensemble. Le président de la République, on a fait une proposition pendant la campagne présidentielle, je le sais bien roule avoir lourdement poussé. Nous avons des marges d'amélioration en cours via le recours au droit souple et par des Côtes d'entreprises comme le code Afep-Medef que vous connaissez et qui fait quand même autorité. Vous dire que nous avons des perspectives assez positif pour. Mettre en place au sein du code Afep-Medef, dans le cas d'un droit souple une corrélation possible entre la performance extra-financière et la rémunération du dirigeant. Il va falloir qu'on soit assez vigilant et qu'on suive cette évolution du code AFEP mais MEDEF je vous cache pas, notamment sur l'intégration d'un ou plusieurs critères environnementaux et sociaux et des critères quantitatifs, qui vont devoir être privilégiée mais l'engagement du MEDEF et de l'AFEP et déjà plutôt favorable par le truchement du droit sous pour faire évoluer la rémunération des dirigeants à l'aune de la performance extra-financière je ne manquerais pas, dès que j'en saurai plus de vous de réunir informer, je vous remercie. Vous souhaitez la réplique monsieur le Lemoine. Très bien merci. La parole est à monsieur Rémy Cardon. Pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Madame la présidente, madame la Ministre, chers collègues, je sais bien évidement commencer mon propos en remerciant les collègues sénateurs et ayant oeuvré à la réalisation de ce rapport. Si des propositions ne sont particulièrement pertinentes, voire même pour certaines trivial. Je pense notamment à la différence de traitement pour les TPE et d'autres me semble sujet à débat. Débat que j'ai donc le plaisir de, d'ouvrir. Pour mon groupe pour lequel j'espère. Que nous aurons des échanges enrichissants. Car le rapport le montre bien, l'ARS est un sujet complexe et sur certains aspects paradoxal. Ainsi d'un. D'un côté la RSE souffre d'une déferlante de des normes qui inquiète, notamment les PME de l'autre côté. Est encore un fourre-tout. Malgré ces normes justement en effet derrière la RSE. Nous pouvons retrouver. La 5 conformité à des référentiels ou à des normes de qualité, on avait envie de formation de fondation pour financer ses projets sociaux et culturels et et j'en passe. Les politiques sociales particulières m'a engagée avec l'ensemble des des congés en réalité de plusieurs mois comme n'oserait à peine l'espérer certains mouvements féministes. respon, la responsabilité sociale des entreprises est défini par la Commission européenne comme l'intégration volontaire j'insiste. Volontairement sur le mot volontaire. Volontaire par les justement les entreprises de préoccupations sociales et environnementales. À leurs activités commerciales et. À leurs relations avec les parties prenantes. Le Champ des possibles est encore immense. Et si les normes sont déjà nombreuses pour imposer cette démarche volontaire, il reste des zones libres, pour ne pas dire de non-droit. la fenêtre d'inévitables inégalités entre les entreprises. Une proposition que j'aurais personnellement aimé voir plus haut dans la liste puisqu'elle arrive en dernier, c'est la modification du du code des marchés publics. Il est évident que les entreprises qui s'engagent volontairement dans une démarche vertueuse et socialement bénéfique et durable. Elle devait être reconnu et engagé pour cela nous arrivons là sur une notion d'exemplarité de l'État qui doit par un code des marchés publics moderniser et favoriser les candidats vertueux. l'expérience montre malheureusement que si on attend que les entreprises s'y mettent spontanément on peut attendre longtemps. Et qui aurait pu prédire que le non partage des superprofits se transformerait en super dividende. Madame la ni sur ce sujet, il est encore temps d'agir. Ensuite, et s'en remettent en cause des propositions qui seront faites puisque la production des chiffres extra-financiers tend à se développer et qu'il s'agit d'une opportunité à saisir. Je trouve que nous devrions nous interroger sur l'intérêt et la pertinence même de la RSE et aux inégalités qui peut engendrer entre les entreprises de différentes tailles. Il est facile en effet pour les grands groupes internationaux de financer une politique. RSE. Généreuse quand ils se sont de fait. Extrait de leur responsabilité sociétale en pratiquant une optimisation fiscale. Mais la première contribution sociétal. Une entreprise n'est-elle pas de participer à la mise en place des services publics aux infrastructures de transports, services de santé et autres services régaliens. Pour le dire autrement. Est-ce la place de l'entreprise de financer directement des services sociaux à l'attention de ses seuls salariés ou à l'État d'en assurer son juste équilibre pour l'ensemble du pays. Madame le ministre à l'heure où nous cherchons à équilibrer le financement de nos retraites, une fiscalité plus juste et surtout plus effective. Quelle que soit la taille de l'entreprise ne serait-elle pas souhaitable. Ce serait de plus. Bien plus acceptable socialement. Et nous vous éviterez les grèves à venir mais ça c'est votre choix. Enfin pour prendre une, une des propositions du rapport que j'ai déjà évoqué. La modification du des marchés publics. Je pense qu'il faudrait aussi intégrer une contribution fiscale des entreprises ainsi les les PE qui qui sont bien souvent ne peuvent pas justement optimisée à outrance, leur fiscalité aurait une bien meilleure note que les grands groupes qui, eux, use de cette optimisation car. De nombreux exemples ont montré l'incapacité du du RSE avec une recherche de revenus à court terme des entreprises. L'exemple le plus marquant en la matière et quand même de mon point de vue le limogeage du président du de Danone dans la politique pourtant exemplaire n'était pas au goût des actionnaires. Ainsi les meilleurs Politiker et se. Souvent avant tout les intérêts de ces entreprises au détriment d'un intérêt commun et supérieur. Madame le ministre, il n'y a-t-il pas de danger a laissé ses entreprises financer ces services sociaux supra légaux au détriment du plus grand nombre pour conclure plus. Je souhaite que le gouvernement reprenne les les propositions bienvenue du rapport et en profite pour prendre encore plus de recul et s'interroge justement sur la philosophie sur le bien-fondé ses limites de la RSE. Je vous remercie. Si cher collègue Madame la Ministre, vous avez la parole. Monsieur le sénateur, votre. Intervention. Est intéressante et étayée par rapport à l'histoire de la responsabilité sociale de nos entreprises. Fut un temps, mais vous devez être plus jeune que moi ou dans les années 2000, on parlait de développement durable. Hou là. Véritablement. Chaque entreprise, peu importe sa taille. Faisaient un peu ce que bon lui semblait communiqué d'ailleurs ne prenait pas beaucoup de risques puisqu'il y avait assez peu de vérifications. Ça faisait des beaux rapports annuels. Mais ça non je ne changeait pas véritablement la vie des entreprises. Et puis en 2014. Les choses sont devenues un petit peu plus sérieuses, vous le savez avec. La des PUF, déclaration de performance extra-financière qui. En anglais, nfr des la non-Finance sur le reporting directive a quand même elle commencer à. À orienter pour toutes nos entre les entreprises européennes de plus de 500 salariés. Des informations relatives aux questions environnementales aux questions sociales de personnel et au respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption. C'était donc je me permets de reprendre votre expression depuis à peu près, bientôt 10 ans, déjà un peu moins fourre-tout. Et puis moi j'ai le sentiment que Postes NF Ferdi arrive c'est SRD alors que nos grandes entreprises, les grandes entreprises ont huit ans de pratique de déclaration de performance extra-financière à partir de critères. Assez exhaustif mais ces critères, ils ont un problème et on s'en reparlera c'est que ils étaient variable une entreprise à l'autre et c'était. Un peu en fonction des, des envies de chaque entreprise. La grande révolution et je pèse mes mots de CSR des. C'est quand même de travailler à partir des mêmes indicateurs et donc de pouvoir enfin comparer la performance extra-financière environnementale, sociale et de gouvernance des entreprises à partir des mêmes indicateurs. C'est vraiment le, l'enjeu de CSR des de pouvoir comparer à partir d'indicateurs convergents. Et je veux quand même rappeler qu'il y aura. Non plus 130 mais plutôt 80 indicateur qui vont, qui doivent permettent de comparer. à dire que je ne suis pas favorable au fait que les entreprises puissent aussi communiquer plus spécifiquement sur certains indicateurs qui sont très en lien avec leur politique sociale ou environnementale, ça ne me choque pas. Donc c'est posent qui met en place des indicateurs et une liberté laissée à l'entreprise aussi de communiquer et de faire savoir ce qu'elle souhaite mettre en avant, plus particulièrement, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait d'opposition pour vous répondre, je suis un peu trop longue entre la RSE et et l'extra-financier. Je pense que l'extra-financier est enfant de l'ARS. Ce qui est d'elles-mêmes en font du développement durable. Je vous remercie. Merci, madame la Ministre. Monsieur vous souhaitez utiliser votre réplique. Merci madame la présidente. D'être rebondir sur la. Le. Les propos de madame la ministre. Je vous. Après tout, votre gouvernement a bien choisi de. Je prends un exemple très concret dans mon territoire, votre gouvernement a bien choisi de décerner le le le prix tschüss France à la société Procter et Gamble à Amiens. Et ce malgré le fait que ces dernières pratiques ne notoire. Fait une sacrée optimisation fiscale contestable et ces derniers légalement totalement. Amoral je dirais prive les salariés d'une juste prime d'intéressement et de participation. Vous voyez un peu le le le décalage entre la remise d'un prix et la réalité. Pour les salariés. Malheureusement. Voilà c'est c'est la, la déception et ça doit être là encore une subtilité du en même temps macronien qui échappe à appeler à la partage de la valeur tout en laissant les entreprises faire le contraire. Merci, cher collègue, la parole est à madame Céline Brulin, pour le groupe CRCE. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. D'abord merci au rapporteur de la délégation aux entreprises pour leur travail qui met en lumière les conséquences de l'application de nouvelles normes environnementales, sociales ou de gouvernance sur nos entreprises et en particulier vis-à-vis des autres pays européens. Il pointe à un grand décalage, me semble-t-il entre les discours et les actes entre les objectifs définis et les politiques adoptées le rapport illustre par exemple que la France est particulièrement mal classé dans le rapport mondial sur le développement durable en raison de son niveau élevé d'importations. Celles-ci représentent la moitié des émissions nationales dans le bilan carbone de notre pays agir efficacement pour des relocalisations industrielles comme dans le secteur de l'industrie pharmaceutique par exemple alors que nous sommes dans un état d'hyper-dépendance aux économies du Sud-Est asiatique notamment à apparaît donc de ce point de vue là aussi une nécessité de même en 2017, la France a été la première avec la loi sur le devoir de vigilance à définir la responsabilité des entreprises et à prévenir les atteintes graves envers les droits humains et l'environnement dans leurs chaînes d'approvisionnement. Mais la directive de voir de Vélizy lance approuvé par le Conseil européen en décembre dernier n'inclut ni l'usage qui est fait des produits commercialisés par les entreprises, ni les activités des clients des entreprises de service, ni même les exportations d'armes sous la pression de la France, les banques sont quasiment exclus du Champ et les entreprises ne sont pas tenus de cesser leurs relations avec un fournisseur qui viole les droits humains, si cela est préjudiciable à leur activité. Il est urgent d'encadrer de façon stricte, l'activité la responsabilité sociale, économique et environnementale des entreprises multinationales et le rapport de la délégation aux entreprises présente plusieurs recommandations intéressantes celle visant à renforcer la formation des membres des conseils d'administration et comité de direction par exemple ou l'instauration de modules de formation sur les enjeux de RSE pour les étudiants ou encore celle sur la progressivité pour ne citer que celles-ci, une responsabilité sociale, sociétale des entreprises, qui ne doit pas se limiter à la seule lutte contre le réchauffement climatique mais inclure les aspects sociaux sociaux ou de gouvernance des entreprises pour mieux devenir une responsabilité sociale des entreprises. À l'opposé des ordonnances Macron qui ont affaibli les pouvoirs de des représentants des salariés dans les entreprises. La consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques de l'entreprise devrait à nos yeux, devenir une obligation. Les salariés pourraient ainsi par exemple s'opposer à des décisions de délocalisation, contraire à l'intérêt général ou promouvoir des diversifications de production à même de développer les entreprises, j'ai en tête par exemple l'équipementier Compin dans l'heure qui délocalisent des productions licencie. La moitié des salariés du site d'Evreux, alors même qu'il s'est engagé à le mobilisé pour équiper le matériel, le matériel ferroviaire financée par la région Normandie. Enfin de mieux valoriser les démarches RSE des entreprises l'introduction dans le code de la commande publique d'un droit de préférence pour les offres des entreprises présentant des atouts en en la matière, à égalité de prix oui équivalente d'offres apparaît judicieux. L'accès aux appels d'offres des PME locales doit en effet être une priorité. Cela demande de cesser de promouvoir des collectivités XXL qui surenchérissent les niveaux d'appel d'offres des groupements hospitaliers toujours plus gigantesques qui éloigne d'autant TPE et PME de la réponse à ces appels d'offres au contraire considérer la politique sociale et environnementale des entreprises peut permettre de dépasser les logiques de dumping social. Nombre de collectivités sont prêtes à jouer pleinement ce rôle mais elles-mêmes soumises aux règles européennes de concurrence prétendu libre et non faussée sont empêchés d'utiliser comme elle le devrait le levier de la commande publique les toi l'état pardon doit également donner l'exemple en la matière et ça, ça n'est malheureusement pas toujours le cas. L'État actionnaire d'abord, je pense notamment à l'l'entreprise Renault particulièrement implanté dans mon département de Seine-Maritime où il accompagne la stratégie de démantèlement qui menace employes sites industriels est nécessaire transition énergétique. Je pense aussi à l'État tout court. Si vous m'autorisez à le dire ainsi se féliciter que les TPE accède à l'énergie a un coût de 280 euros le mégawattheure, c'est-à-dire 5 à 6 fois supérieur au coût de production en France n'est pas très sérieux. Vous le savez, nous sommes évidemment diamétralement opposées à Milton Friedman qui considéraient que l'entreprise a pour seule responsabilité d'accroître son profit mais à l'inverse, nous considérons que l'état la puissance publique ont aujourd'hui une responsabilité à l'égard de toutes nos entreprises face au coût de l'énergie et que les réponses apportées à ce stade par le gouvernement ne sont Madame la Ministre pages à la hauteur. Vous avez parlé d'urgence. C'est je crois le sujet particulièrement urgents qui les préoccupent aujourd'hui je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. C'est une ironie du sort ou pas mais. Compte tenu du fait qu'il y a eu des petits problèmes pour le vote au Parlement, j'avais le choix. Entre honorer ma présence au Sénat ce soir comme c'était prévu ou porter le débat sur les aides énergie devant les députés. On ne va pas tout mélanger. Je ne vais pas vous répondre sur les aides énergie si j'aurai à coeur de le faire si vous le souhaitez. Dès demain, évidemment vous l'avez dit, nous sommes diamétralement opposées et j'aurai à coeur d'y revenir parce que les 280 euros le mégawattheure lissé sur l'année. J'aurai à coeur de les défendre mais ça fera l'objet d'un autre débat. Deux 3 choses. Vous avez dit beaucoup de choses dans votre intervention donc je vais aller vite hein. Sur l'empreinte carbone les importations, vous avez raison trois fois raison c'est pour ça d'ailleurs que Bruno Lemaire d'ici quelques semaines voire un mois ou 2 orages je crois le loisir de vous présenter un projet de loi robuste sur la réindustrialisation verte vous m'accorderez que la meilleure façon de faire baisser le bilan carbone de nos importations, c'est de créer les conditions d'une réindustrialisation forte et verte dans notre pays, ce sera l'objet d'un projet de loi qui vous sera présenté dans les semaines et mois qui viennent sur le devoir de vigilance, madame la sénatrice brûlant rappeler quand même que la France est moteur d'autant plus que je n'y suis absolument pour rien puisque c'est la loi. Du député Potier en 2017 qui a fait avancer la France et qui fait avancer l'Europe aujourd'hui rappeler quand même que les Allemands ont emboîté le pas des Français. Et rappelons quand même que l'Europe est aujourd'hui en train de, de porter le devoir de vigilance à partir de l'influence française et d'une France qui a été absolument moteur en la matière, quitte à vous étonner mais j'aime bien être étonnante, si je suis pas très éloigné de ce vous dites sur le CSE et nous pourrions en reparler parce que je crois que si on veut vraiment que l'extra-financier soit incarné et vivent dans nos entreprises et que l'empreinte sociale environnementale et gouvernance soit responsable. Bah, il me semblerait important que les salariés à un moment ou à un autre en soient vraiment parties prenantes je t'ai pas en allant aussi loin que vous mais je trouve que votre intervention sur le CSE est intéressante et si vous l'acceptez qu'on n'en reparle vous avez abordé aussi le sujet des marchés publics. Un sujet majeur sur lequel il me reste plus de temps mais je vais vous dire qu'à l'article 35 de la loi climat et résilience, sur laquelle je me suis engagé ce sujet avait été abordé. Rappelez-vous le Conseil d'État nous avait retoqué sur l'offre écologiquement la plus intéressante. Nous sommes ici encadrée par le droit européen et je vous rappelle que nous avons été repris par le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi climat et résilience, il n'est pas possible en droit européen de promouvoir la notion d'offre écologiquement la plus avantageuse. Vaste ce sujet auquel je travaille depuis des années, reparlons-en avec plaisir madame la sénatrice. Pardon, madame la présidente. Madame Françoise Férat. Pour le groupe Union centriste, chers collègues. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à féliciter la délégation des entreprises pour la qualité des travaux entrepris dans ce second rapport sur la responsabilité sociétale des entreprises, et notamment l'investissement de son président, Serge Babary. Ainsi que celui de nos rapporteurs Martine Berthet Florence d'. Compta et Jacques Le Nay. Plus Khan n'est plus qu'un acronyme la RSE, est désormais au coeur de la vie de nos entreprises. Pratiques de management exigences comptables ou encore transparence des données aucun pan de la vie d'une entreprise n'y échappe. Si les plus importants de nos sociétés n'ont pas de difficultés à se faire servir de ce sujet. Ce n'est pas le cas pour nous ETI et PME qui n'ont bien souvent pas les moyens humains ou financiers pour mettre en oeuvre des stratégies RSE ambitieuse. Pourtant, cette mise en oeuvre revêt une importance déterminante tant pour notre planète que pour la compétitivité des entreprises. Le défi de la transition écologique et de l'adaptation au changement climatique ne doit pas être uniquement d'affaire des collectivités locales, il doit concerner les habitants et les entreprises. Ces dernières détiennent un véritable pouvoir de changement de comportement des consommateurs en proposant des biens et services durables conçu dans une responsabilité sociétale. Souvent en économie et en marketing, l'offre crée la demande. Proposer des produits responsables et qualitatif, ils trouveront preneurs des consommateurs sont très attentifs aux engagements sociaux et environnementaux. Les entreprises. La disparition de la taxe professionnelle et l'annonce de la suppression de la CVAE. Pourrait distendre les Liens entre le territoire et les entreprises. La RS se permette de retisser ce lien. Les plus petites entreprises auront d'ailleurs tendance à avoir un lien de proximité externes à leur taille pour témoigner d'une d'une implication sociétale avec l'école du village ou du quartier. La commune ou des associations locales. La norme ISO 26.000 standard international qui définit le périmètre de la RSE autour de cette thématique centrale prévoit des obligations en matière de communautés et de développement local. Afin de faire de la RS. Un véritable atout pour nos entreprises, y compris les plus petites. Il est donc urgent d'agir, a-t-il à triple titre. Premièrement, mettre en oeuvre un choc de simplification en matière de RSE. Afin que chacune puisse respecter ses obligations françaises et européennes. Notamment dans le cadre de la future directive

Car 2 des 3 piliers de SG à savoir la mise en oeuvre une politique sociale et l'existence d'une gouvernance transparente. Évolue évolue aujourd'hui dans l'ombre de la lutte contre le réchauffement climatique. Et ce n'est pas une responsabilité environnementale des entreprises mais une responsabilité sociétale de celle-ci. Enfin, les pouvoirs publics doivent davantage prendre leur part afin de rendre la RSE opérante. L'obligation d'une clause environnementale dans les marchés publics. 2025 est une première étape. Cependant nous devons aller plus loin. À ce titre je salue la proposition des rapporteurs d'intégrer un doigt d'un droit de préférence. Pour les offres des entreprises ayant une stratégie RSE à égalité de prix ouais équivalence d'offre a-t-elle droit sur un outil précieux pour faire de la RSE, un atout pour la compétitivité de notre prise. Vous l'avez compris, mes chers collègues, si avec les membres de mon groupe. Nous saluons la montée en puissance de l'ARS au sein de nos entreprises vous estimant qu'elle doit être accessible à l'ensemble. Nous devons continuer de travailler pour faire de ce principe une véritable réalité sur le terrain. Et un outil pour la compétitivité des entreprises les plus vertueuses ainsi la ARS deviendra un atout pour notre économie il aux entreprises et je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Merci madame la présidente. Vous dire. À quel point le gouvernement être. À deux fondamentaux que vous avez abordé madame la sénatrice la proportionnalité. La progressivité. Et vous l'avez mentionné, notamment à l'endroit de nos entreprises de taille intermédiaire et j'ai à coeur de vous rappeler que la directive c'est SRD qui est entré en en vigueur le 14 décembre dernier. Ah ah et et l'objectif pour la France est désormais de transposer. On se les dit tout à l'heure cette directive au cours de l'année 2023 et en toute autre à cause d'ici juillet 2024. Il n'est pas possible. Par conséquent, de redéfinir le périmètre des entreprises concernées ou de revenir sur le principe des informations à publier. En revanche, durant la présidence française du Conseil de l'Union européenne, le gouvernement a bien veillé. Et j'ai veillé très personnellement à ce que la directive soit proportionnée pour nos entreprises. C'est le cas pour le périmètre, vous le savez, des entreprises concernées puisque les PME qui n'ont pas émis d'actions ou d'obligations sur les marchés réglementés ne sont pas concernés. En outre, les PME cotées seront exemptés de toute obligation si elles sont couvertes par le rapport de durabilité de leur société mère. Par ailleurs, dans le cas de la consultation sur les. Projet d'indicateurs de reportage. La France sera particulièrement attentive au nécessaire respect de la confidentialité d'un certain nombre d'informations. La directive permet d'ailleurs aux États membres d'autoriser les entreprises à ne pas publier comme vous le savez certaines informations dans des cas exceptionnels, dument. Lorsque ça nuirait gravement à la position commerciale de l'entreprise face à ses concurrents. C'est important de le rappeler. Je veux aussi vous rappeler au-delà de la proportionnalité la progressivité 2025 seront concernés, les grandes entreprises de plus de 500 salariés, coté sur le marché ou exerçant dans les secteurs de la banque et de l'assurance. 2026 les grandes entreprises. 250 500 salariés, 2027 les PME cotées. Avec possibilité de report d'une année 2029 les filiales et succursales de grandes entreprises extra- européenne, nous y avons donc veiller tout particulièrement et pour ce qui concerne les PME, même si ça ne nous empêche pas de travailler et de ne pas ça et ça n'est pas l'idée de de pantoufler de ne rien faire jusqu'en 2027 mais nous avons 5 années devant nous pour les accompagner les prévenir et surtout ne pas faire peur à des PME, ce que vous ne faites pas mais d'autres le font, qui ne serait pas concerné par le Champ de la directive, je vous remercie. Merci, madame la Ministre, la parole est à monsieur Henri Cabanel pour le groupe RDSE. madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues. Responsabilité sociétale des entreprises RSE. Pour les initiés ou comment assumer sa responsabilité face à la société. C'est le mérite d'être connu, la norme ISO 26.000, publié en 2010, apporté un consensus à la RSE. 5 ans de travail pour 99 pays qui ont planché dessus pourtant sa notoriété laisse à désirer. Dans une enquête destinée au maire de mon département 39% des élus ne savent pas ce que c'est que la responsabilité sociétale des entreprises. Sur 17 étudiants en master de, de droit rencontré cette semaine Sam pour ça ne savait pas quels âges l'. 12 ans après, il est donc primordial d'enfoncer le clou. La délégation aux entreprises de à Paris il y a 2 ans du sujet avec un rapport de loterie titré sans ambiguïté une exemplarité à mieux encourager car il s'agit bien de cela, l'exemplarité, que ce soit dans la gouvernance dans le respect des droits de l'homme dans les conditions de travail dans la contribution au développement local du consommateur dans la protection du consommateur pardon et évidemment de l'environnement. D'abord destiné aux grandes entreprises, l'air et ce s'est adapté et s'est ouverte aux PME et ETI avec une évaluation. Sur 5 principes au lieu de sept. Les enjeux sont hein durant le manteau sociétaux économiques collant au triptyque du développement durable. Dans ce rapport, la délégation des entreprises et présente à des réalités. Un monde qui n'est pas celui des bisounours s'certains ont détourné les enjeux éthiques en affichant une image avant les actes voir ça les actes Green washing ou pour peu soit Chine la manipulation reste la même, en profite de la vague des bonnes intentions pour surfer sur ces, sur le fond. Dans un contexte d'après-Covic de, de vide et de crise économique, énergétique. Certaines entreprises ont démissionné du processus. D'autres se sont désengagés ou ont baissé la garde général leur expulsion de la labellisation certaines. Du coup, critique ce qui ce qui les avaient pourtant motivé là je. L'image est primordial dans un contexte de concurrence mondiale et donné dénigrement du Label est une revanche pas très pas très fair-play pour des groupes qui s'sur le service à la limite dans leur stratégie de communication. C'est précisément ce contexte de concurrence mondiale qui doit pousser la France et l'Europe à défendre la norme ISO 26.000 qu'il faut réaffirmer plutôt d'ailleurs que reporting qui ne fait que référence à aucune non Les experts savent que les Américains qui ne partagent pas les mêmes valeurs de l'entreprise ont toujours voté contre et qu'ils ont créé bicore une norme moins robuste et moins crédible. Concrètement. Pas d'évaluation sur chiites et pas d'écoute dans les parties prenantes externes et internes. Un vrai chant des sirènes pour certaines entreprises qui se disent qu'elles bénéficieront de l'image de la labellisation c'est gros ce compte Print. Et c'est là tout le danger d'un j'ai encore concernant l'espionnage qui s'organise via des structures d'évaluation étrangère. L'Europe doit défendre sa vision humaniste éthique et environnemental de l'entreprise. Il y a donc, comme le souligne ce rapport une nécessité accompagner les petites entreprises à la prise en compte de la RSE. Incontournable dans les cinq ans. Mais cela doit se faire dans le respect des textes fondateurs que sont le. RD et la norme ISO 26.000, le CHRD publié au JO de l'Union européenne depuis le 1er janvier et qui devra être rapidement a piqué en France. Elle précise le nouveau cadre européenne de reporting de durabilité. Concernant la norme ISO 26.000. Rappelons qu'elle est le seul guide méthodologique reconnue internationalement. Il est souvent question de reporting mais cela n'était pas une fin en soi. Ce qu'il faut soutenir c'est la RSE dans la stratégie d'organisation des structures le reporting ça va ça vient après. Plus simplement dit ce n'est pas l'outil qui fait l'artisan. Fait je ne manquerai pas l'occasion de ce débat. Pour vous donner un scoop, madame la Ministre, mon cabinet viennent de recevoir hier l'attestation la engagé RSE ce niveau exemplaire que nous avions eu déjà à 2019. Mon cabinet toujours le seul en France à être labellisé ma directrice de cabinet et mon attachée parlementaire que je tiens à remercier publiquement porte avec motivation et détermination, cet engagement dans mes côtés. Stratégie demanda télétravail. Et covoiturage avant que ce soit à la mode comptabilité avant que ce soit obligatoire. Indicateurs de résultats etc. Une simple méthode sans usine agace. Je remercie également l'Afnor Certification qui nous a fait confiance à 2015, quand nous leur avions indiqué notre intention d'engagement mon projet, créer la responsabilité sociétale des élus. 72. Héraultais m'ont déjà affirmé leur intention de participer à un groupe de travail que j'ai initié une force à mes côtés, je vous rappelle que nos cabinets on tous un numéro Siret et que nous pouvons donc nous engager. Ce. Car mes chers collègues. Qui mieux que nous. Dans ce contexte de défiance. Devrait s'engager face aux citoyens. Ne pouvons-nous pas être exemplaire comme nous demandons aux entreprises nous leur imposons des obligations toujours plus lourde c'est facile pour les autres mais plus compliqué pour soi-même. C'est pourtant le sens même de l'exemplarité montrer l'exemple. Le défi est lancé. Je vous remercie. Chiche, Monsieur le Sénateur Cabanel parce que. D'abord je trouverais très intéressant si vous acceptiez qu'on partage. La labélisation que vous avez reçu. Je suis très sensible à ce que vous avez dit sur l'exemple. Et a priori plutôt favorable même si je pense qu'ici il y a quand même plutôt des élus. Responsables. Ceci est allemand et engagé. Je pense que c'est au coeur. De notre fonction d'élu. Mais je trouve l'initiative particulièrement pertinente, c'est pas un mot en l'air. Si on a l'occasion d'en reparler. J'aimerais bien qu'on en reparle parce que ça m'intéresse. 3 petites choses, vous avez mentionné les étudiants. C'est même très intéressant. Vous me dites 100% des étudiants du master. Et 80% des étudiants du master ne savent pas ce qu'est la responsabilité sociale des entreprises ou ce que ça recouvre. Et en parallèle, vous avez de plus en plus de Chair de master de formations, qu'elle soit, continue d'ailleurs ou ou secondaires sur ces enjeux et même des écoles aujourd'hui dans des instituts prestigieux français sur l'impact. donc ça se déploie. Est-ce que ça se déploie pas assez sur les formations plus classique universitaire sujet important que d'ailleurs les sénateurs et sénatrices ont mentionné dans le rapport et auquel je j'adhère totalement. Mais il y a quand même de plus en plus de formation aujourd'hui pour embarquer notre jeunesse qui est très désireux, sur ces enjeux de RSE. La RSE et vous le savez aussi, c'est un peu Monsieur Jourdain. Il y a beaucoup d'entreprises qui la pratiquent, sans forcément le savoir et notamment nos plus petite. Quand un directeur de PME de TPE a fait du partage de la valeur des actions gratuites. À une politique associative. Suivi, il ne sait pas forcément que ça s'appelle. De l'extra financiers ou du développement durable la responsabilité sociale et pour autant son nez. Je suis en revanche. Pas d'accord sur un point, je crois que pour le coup outil va cher l'artisan. Je crois qu'il est indispensable qu'on avance ensemble sur ces ensemble en Europe. Sur ces 80 macro-indicateurs qui sont transe sectorielles comme vous le savez avant d'enclencher un travail plus sectorielle en fonction des secteurs d'activité, mais je pense qu'il est indispensable que l'outil même s'il est un peu lourd et qu'il faut l'adapter aux PME. Soit homogène pour que justement nous parlions le même langage. Ça fait 20 ans que je suis passionné par ces sujets, et 20 ans que je me désole parfois qu'on compare des choux, des carottes, des tomates avec des politiques sociales et conclut très différents dans les entreprises. L'outil est indispensable. J'espère qu'il fera l'artisan d'une RSE MEG dans les entreprises. Merci. Monsieur Cabanel. Merci madame la présidente. Madame la mi-mai ministre oui vous l'avez bien. Dit l'outil fait pas l'artisan mais. Vous avez raison. L'outil est indispensable mais. Il était important d'avoir la philosophie aussi pour s'engager et je le sais très bien moi. Qui agriculteur monsieur engagées en bio. Je sais qu'il y en a qui ont profité donc de cet engagement par rapport à des, des retombées financières. Je pense qu'il faut la philosophie et dans ce cadre de la RSE. C'est exactement pareil, il faut vraiment la philosophie concernant la RSI et bien entendu Madame la Ministre je reste à votre disposition. Merci, cher collègue, la parole est à monsieur Stéphane Sautarel pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente, madame la ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs. Je veux d'abord saluer le travail de la délégation aux entreprises du sénat autour de la responsabilité sociale des entreprises sociétal pardon des entreprises travaillent inscrit dans la durée, sous l'impulsion de son président, Serge Babary. La RSE doit être à la portée de toutes les entreprises nécessitant une adaptation des exigences à l'échelle de chacune et dans un cadre européen. En ce sens je souscrit aux propositions de la délégation aux entreprises. Mais la RSE, c'est aussi et d'abord une question de culture, d'état d'esprit avec un rôle essentiel des conseils d'administration qui confère à l'entreprise un rôle nouveau d'intérêt général. Je veux donc profiter de ce temps pour élargir le débat tout en m'inscrivant je le crois. Au coeur de celui-ci. La RSE. C'est d'abord la sincérité et l'exemplarité. Au delà de la sincérité du dirigeant qui ne peut s'ancrer que dans la durée et dans l'exemplarité. Le cadre collectif, le cadre juridique peut aussi aider à poser cette sincérité cette ambition. C'est ainsi que la RSE s'inscrit dans le dépassement de l'entité à la fois en direction de l'intérêt collectif qui la transcende et d'une attention individuelle réelle et sincère qu'il habite. La RSE, est un moyen de s'engager de manière forte et sincère. Avec des tiers certificateur garantissant cet engagement cette intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leur activité commerciale constitue une réelle avancée. À l'occasion de la préparation de la loi pacte Nicole Notat et Jean-Dominique Senard ont produit un rapport relatif à l'entreprise. D'intérêt collectif. Ils ont ainsi conduit une mission sur la relation entre l'entreprise et là as entre Le rapport qui avait vocation à être prises en compte dans l'élaboration de la loi pacte présente un intérêt certain pour asseoir la légitimité l'authenticité, la sincérité, indispensable à l'émergence d'une telle approche qui peut être qualifié d'humaniste. La loi pacte qui ambitionnait de donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer de grandir et de créer des emplois n'a pas encore donné toute sa mesure et mériterait une évaluation de dynamique d'envergure tant sa portée considérable. Je suis sûre Madame la Ministre que vous partagez cet enjeu et cet objectif. Elle a posé le fait que l'entreprise poursuivent un 2ème objectif parallèlement à sa profitabilité sa raison d'être la raison d'être peut se définir par l'expression d'un futur désirable pour le collectif partie constituante et prenante justifiant la coopération et rendant compte d'un enjeu d'innovation cette raison d'être but propres de l'entreprise en tant que personne morale, pourrait permettre de renforcer l'engagement des salariés en étant porteur de sens. La réappropriation par l'entreprise de sa responsabilité comme d'une raison d'être associé à une officialisation stratégique voire juridique apparaissent être de bonne piste. La responsabilité sociale, sociétale est ainsi décryptée à travers 3 niveaux d'engagement la considération des impacts sociaux et environnementaux liés à son activité. La réflexion sur son environnement à long terme et enfin le statut de société à mission. Longtemps considérée comme contribuant au problème. Nombre d'entreprises souhaitent aujourd'hui faire partie de la solution. Ces défis écologiques, sociaux scientifiques de plus en plus d'entrepreneurs ambitionne de les relever à travers l'entreprise il y a là une opportunité historique historique d'ouvrir la voie à de nouvelles formes d'entreprises qui pourrait bien dessiner les contours d'un capitalisme du XXIe siècle passant l'intérêt des humains et de la planète au coeur de ses finalités intégrant de nouveaux modes de partage de la valeur créée. À cet égard, l'évaluation de la RSE mais aussi de la mise en oeuvre de la raison d'être par un tiers, indépendant et la reddition publique par les organes de gouvernance est une nécessité absolue. La loi doit aider les entreprises à placer au coeur de leur projet. La résolution des enjeux de société, sociaux et environnementaux. Elle doit aider à crédibiliser la démarche. Les pouvoirs publics pourraient ainsi transférer ou partager avec l'entreprise, la définition de l'intérêt général pour la société mettant le chef d'entreprise, c'est-à-dire les organes dirigeants au coeur d'une mission politique et historique, ce serait un changement radical de l'organisation française. Ainsi, on pourrait espérer que l'époque ne soit plus à la défiance mais à la confiance. Assis sur la sincérité des engagements et des convictions, il apparaît que cette approche peut et doit permettre de faire que la performance durable devienne excellence la sincérité et première dans cette démarche. C'est pourquoi les 5 propositions de la délégation doivent être mises en oeuvre pour franchir une nouvelle étape et j'espère Madame la Ministre que vous pourrez à votre niveau, prendre en compte ces propositions, je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Je. N'ai pas véritablement de de de. Question, mais je tiens à revenir sur. Ce que vous avez dit monsieur le sénateur sur la loi pacte. Il est des lois qu'on présume qu'on oublie pas voter à 5h 12 du matin le 22 mai 2019. Et donc vous connaissez mieux que moi le temps du Parlement. 19 plus 3, le temps de l'évaluation et peut être venu, et vous me trouverez toujours à vos côtés pour. L'évaluer. Et peut être la renforcer l'améliorer. Vous dire aussi que je n'ai pas attendu les trois ans. De coutume pour continuer à faire avancer cette loi notamment son chapitre 3 et. Comme vous l'avez rappelé le le travail sur les sociétés à mission la raison d'être. Vous avez beaucoup utilisé de sincérité Monsieur le Sénateur, je suis très sensible. La sincérité. C'est comme la confiance, ça n'exclut pas le contrôle. Vous dire que j'avais aussi missionné Brice Rocher, vous vous en souvenez sûrement, les sénateurs et sénatrices de la délégation, le ça, vous avez mentionné le rapport dans vos travaux. Et vous dire qu'il y a au coeur des travaux de Brice Rocher des propositions plutôt plutôt pertinentes dont certaines sont soutenues par le rapport de la délégation vous donner une explication sur le pourquoi. Parce que je suis plutôt en général. Assez réactive sur ces enjeux, sur la société a mission mais on a été frappé de plein fouet par la crise Covid. Ce qui a empêché. Toute une première vague de bilan de rapport que les organisations tiers indépendante qui viennent contrôler la qualité de la mission annoncé par l'entreprise n'ont pas pu remettre en temps et en heure, donc les premières sociétés mission vous le savez, sont des dès 2020 des même la fin d'année 2019 et on commence tout juste à avoir les rapports des OTI sur l'émission et leur adéquation avec le coeur de métier de l'entreprise. Un sujet que vous avez aussi abordé le fait que la mission était parfois un peu éloigné du coeur d'activité de l'entreprise et je pense que d'ici quelques semaines. À mon avis, très peu de moi, on va avoir beaucoup plus de rapports d'OTI permettant de qualifier. Et donc d'améliorer peut-être la sincérité de la mission comme de la raison d'être pour ce qui est de l'intégration de la raison d'être dans les statuts. Je suis acquise. Totalement acquise à cette idée, je vous remercie. La parole est à monsieur Emmanuel Capus pour le groupe les indépendants. Merci madame la présidente, madame la Ministre, mes chers collègues. La notion de responsabilité sociétale des entreprises est essentiel. Pourtant, force est de constater que la culture RSE. Traverse une période difficile. La crise sanitaire a mis nos entreprises à rude épreuve. Le contexte économique tendu, que nous connaissons et tout particulièrement la hausse des coûts de l'énergie inscrit nos entreprises dans une course d'endurance difficile. Bon nombre de nos entreprises sont inquiète. Au même moment. On l'a entendu une petite musique se fait entendre. La raison d'être des acteurs économiques ne seraient pour certains que de l'esbrouffe destinée à donner une bonne image à des entreprises faussement engagé. Bref, de l'éco-blanchiment ou du porc washing en bon français. Dans ce contexte, le rapport alerte sur le fait que certaines entreprises pourraient être tentées voir forcés. De négliger leurs engagements environnementaux et sociétaux. Pour couronner le tout, la complexification des obligations en matière de de RS. Ne cesse de croître et nous interroge sur leur accessibilité à l'ensemble des entreprises. Ces risques doivent nous mobiliser tant l'ARS bien loin d'être superflue est au contraire un atout majeur pour gagner en compétitivité. L'ARS participe à garantir la vitalité de nos entreprises à pérenniser leur implantation et ainsi à renforcer le tissu économique local. Pour atteindre ces objectifs. Nous devons la revoir d'un oeil neuf. Nous interroger sur l'inflation normative adapter les règles aux enjeux actuels. C'était justement l'objet d'une proposition de notre groupe à la suite de la mission d'information conduite par Vanina Paoli-Gagin il s'agit d'élargir les critères de responsabilité sociétale des grands groupes en incitant leur collaboration avec les Start-Up et PME innovantes. Dans le même sens. Si nous parlons de RSE. Nous ne pouvons oublier une notion développement la RTS responsabilités territoriales des entreprises. Je crois que nous n'avons pas abordé cette question. La RTA permet d'appréhender le territoire d'implantation. Comme un espace d'ancrage responsable d'engagement sur le temps long et de collaboration public-privé. Dans une logique écosystémique la RTE représente un axe fort de valorisation dont témoigne l'enquête des dévoilé, en novembre 2022 par SS France la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Selon elle, les missions prioritaires des entreprises sont la création d'emplois. La prise en compte de la transition écologique et enfin le soutien aux filières locales. L'interdépendance progressive entre les acteurs économiques d'un même territoire ne peut qu'inspirer une approche globale de développement mutuel. Enfin les études montrent que les salariés sont en attente de formation pour participer activement aux engagements de leur entreprise et donner du sens à leur mission quotidienne. Développer l'accès à la formation permet de changer les mentalités et d'atteindre de vrais résultats pour la mobilisation collective à toutes les échelles. Notre rôle est de continuer à bâtir un environnement propice à la bonne bonne santé économique de de nos entreprises. En concrétisant des politiques de RS et de RTE. Elles en sortiront renforcées et pourront contribuer au développement de leur territoire d'implantation. Dès lors, Madame la Ministre j'émets le souhait au nom du groupe les indépendants. Que la notion de territorialité soit davantage pris en compte par les entreprises dans leur activité. Je vous remercie. Merci cher collègue Madame la Ministre. Votre discours monsieur le sénateur, qui a pu ne peut obtenir que mon adhésion totale et et massive, c'est frappé sous le coin du bon sens mais comme il est de bon ton de rappeler le bon sens. Je vous en remercie. Je me disais on vous écoutant mais ça n'empêche pas de le faire. Concomitamment pour éviter en même temps. Tout le combat qu'on mène, et les sénateurs et sénatrices qui ont qui ont porté le rapport le savent et c'est pas rien, c'est 2 et la France a été moteur ça a été d'embarquer quand même ce sujet au plan européen. Pour que dans les 27 États membres et notamment en Europe de l'Est dont la culture, vous avez été nombreux à en parler de la RSE, est très différente de la notre, voire dans certains pays. Naissante voire balbutiante on arrive ensemble et vous l'avez mentionné, ainsi que le sénateur juste avant vous sénateur Cabanel on a. Aujourd'hui, une obligation enfin une obligation une volonté en Europe de faire en sorte. De défendre notre modèle de capitalisme européen. Et les premières interventions revenait sur le devoir de vigilance madame brûlant notamment sur les droits de l'homme sur. Et c'est un combat titanesque, il nous faut mener pour partager. Au-delà de ces indicateurs ces ces ces pratiques d'entreprises dans l'ensemble des pays européens. Au plan environnemental, social et de gouvernance. Donc c'est vrai que comme je suis plutôt dans une dynamique de comment on continue à pousser, nous la France en matière d'exigence l'Europe. C'est vrai que j'ai, j'étais pas déstabiliser mais je trouvais intéressant de vous écouter, vous êtes pas le 1er non plus, je crois que vous aussi, monsieur le sénateur, vous l'avez mentionné, n'oublions pas le local mais d'ailleurs ça ne l'empêche pas donc. Peut être peut-on regarder travailler, il faut que je regarde un peu les indicateurs et que j'y travaille avec le Trésor mais ça me semblerait pas du tout hors sujet de. Pousser peut être ou de travailler sur des indicateurs. Territoriaux une application territoriale dans le cadre d'une performance extra-financière des entreprises se comportent en Europe. Merci. Le bon sens est toujours de bon ton a rappelé donc je, il faut qu'on regarde, je vous remercie. Si Madame la Ministre. La parole est à Madame, Florence. Trix compta. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais tout d'abord remercier le président Serge Babary d'avoir proposé ce débat. Portant sur la proposition de résolution de notre délégation aux entreprises car développer la RSE est important pour pour l'ensemble de nos économies de nos entreprises, bien sûr, mais aussi pour notre économie car notre monde est en pleine mutation. L'effort conséquent que nous devons consentir pour nous y adapter concerne aussi nos entreprises, c'est-à-dire les valeurs qui les fondent les hommes et les femmes qui travaillent les objectifs qu'elle poursuivait les produits qu'elle fabrique aux entreprises en France et en Europe sont confrontés à 3 défis majeurs. Le défi déjà ancien de la compétitivité face à une concurrence internationale toujours plus aiguisé, le défi de la transition énergétique et écologique. Il est fondamental et nécessite d'adapter tout le process de production et de services aux impératifs du changement climatique et enfin le défi du capital humain. Nos entreprises peinent à conserver dans la durée, leur cadre soucieux de plus d'autonomie d'une responsabilité différente elle peine également à attirer les plus jeunes, les meilleurs diplômés par la seule promesse de stabilité professionnelle ou d'une bonne rémunération là encore à la crise sanitaire a rendu tangible à tous. Cette réalité, le bien-être au travail. La quête de sens dans le travail sont aujourd'hui au coeur des problématiques de recrutement dans ce contexte j'ai générale et face à ces 3 défis majeurs. Les entreprises françaises dispose d'atouts solides. La France a été précurseur en matière de RSE. Il s'agit aujourd'hui de conserver ce Leadership et d'en faire un atout pour nos entreprises. Depuis des années maintenant. La RSE ASM a essaimé un peu partout, les grands groupes et entreprises s'en sont saisis et communique beaucoup sur cette démarche. Je m'en réjouis, mais il s'agit de faire plus et mieux. Il ne s'agit plus de dire que l'on fait mais de faire réellement la la RSE doit être partie intégrante du Business model de l'entreprise pour lui conférer des atouts à la mesure de ses engagements. L'accélération normative que nous avons évoqués européenne mais aussi des autorités françaises en ce domaine est très importante. Le ce rapport en rencontre de façon détaillée par exemple depuis le 1er janvier de cette année, les entreprises de plus de 50 salariés réalisant 40 millions de chiffre d'affaires ou 20 millions de total bilan vont devoir réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre particulièrement exigeant la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises que l'on a évoqué la directive CSR dès qui se propose d'harmoniser de standardiser ce reporting est entré en vigueur le 5 janvier dernier, elle élargit considérablement le périmètre à des sociétés entreprises potentiellement soumise à la publication d'informations extra-financière. On estime à plus de 50.000 entreprises européennes, 5 fois plus qu'actuellement et ce Laura. Cela a été dit, un effet sur nombre de PME sous-traitantes ou co-contractante donc ça leur a cela affectera largement notre tissu de

Et ça, nous sommes vraiment souhaitable concernant les PME si le reporting et son contrôle sont essentielles. Il est indispensable d'aller au-delà de ce contrôle faute formelle et d'accompagner réellement les PME dont les finances sont contraintes dans l'évolution de leurs pratiques, elles ont besoin d'être accompagnés. Il me semble aussi important important d'accompagner. Les les les auditeurs des Pays-Bas nous nos petits auditeurs qui n'ont pas les moyens en matière de RSA. Les, les moyens de conseils, notamment des Big Four. pour conclure l'ARS. Oh c'est pas simplement un effet de mode mais un vrai levier au bénéfice des économies et des entreprises européennes pour qu'elle se dote d'un atout majeur. Je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la Ministre. Merci madame la présidente vous répondent peut être à madame la rapporteure d'ores et déjà parce que je l'avais pas fait par le pour le. Le précédent sénateurs ou sénatrices sur. Les professions du chiffre et les commissaires aux comptes, notamment les commissaires aux comptes vont avoir un rôle important dans l'application de la CIA cerné. Ils le savent. La compagnie nationale des commissaires aux comptes la CNCC est déjà très active très en avant sur le volet formation pour former ces professionnels parce que la performance extra-financière fait appel à des compétences nouvelles et donc c'est un chantier qui est en cours et et soyez assurés que je m'en assure. Assez fréquemment. Vous dire aussi que je travaille avec le ministère de la justice. Sur les moyens de faciliter l'accès au stage préparatoire au CAC aux personnes qui seraient des professionnels du développement durable et pas uniquement à des professionnels du chiffre ça pourrait passer par exemple par une admission sur dossier plutôt que par concours, pour aussi. Entre guillemets mixer un peu plus les approches entre professionnels du chiffre et professionnel du développement durable, puisqu'il y a derrière ces chiffres que vont glaner les indicateurs. De la directive CSSD aussi des pratiques en matière environnementale, sociale et de gouvernance qui suppose des connaissances parfois au-delà de la seule comptabilité. Que pratiquent aujourd'hui nos donc c'est un chantier sur lequel nous sommes avec le ministre de la justice avec son ministère et je veux aussi vous répondre. Sur l'Esma que vous avez mentionné l'Autorité européenne des marchés financiers. la France a défendu défend à de nombreuses reprises que soit introduit au niveau européen une réglementation encadrant l'activité des agences de notation. Le sénateur, le Moine laver aussi mentionné et une telle réglementation devrait être proposé par la Commission européenne dans les tout prochains mois. La France suit de très près ce sujet en plus de la directive sur les agences de notation. Je vous remercie. Merci, madame la Ministre, la parole est ta monsieur Jean-Pierre Moga, pour le groupe Union centriste,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues. Je voudrais d'abord remercier comme tout le monde dans le président babary et la délégation aux entreprises d'avoir abordé ce sujet. Si l'on reprend le fil de l'histoire, la responsabilité sociétale des entreprises s'est établi comme CFCM actuel dans le courant des années 2000. D'abord enfin culte hâtive et volontaire. Cette approche méthodologique a permis de fournir une grille d'analyses nouvelles pour la compréhension du rôle des entreprises non non seulement dans le système économique mais plus Gobelins globalement au sein de la société. Ils foutent envisager l'avènement de la RSE comme un contre-pied à la libérer stylisation ainsi qu'à la financiarisation de l'économie opéré à partir des années 80. Ce phénomène. A fini par apporter avec. Lui son lot de questionnements. Quel doit être le rôle des actionnaires dans l'économie. L'investissement notamment privé doit-il poursuivent au d'autre but que la simple rentabilité financière. Les entreprises ont talonne devoir de compenser les externalités négatives liées à leur activité.

La RSE. A dans un 1er temps permis de conceptualiser la manière dont les entreprises ne pouvaient affecter positivement leur écosystème respectif néanmoins. On assiste depuis quelques années, a une influence juridique que croissante de l'ARS. Étant limité par le temps. Je souhaiterais aborder un aspect seuls aspects précis de cette influence. Juridique croissante. L'aime. De la RSE sur le secteur financier a été particulièrement spectaculaire au sein de la décennie qui vient de s'achever, Que l'orientation de l'épargne des entreprises et des ménages vers des activités vertueuse. Sur le plan environnemental ou social constitue indéniablement une avancée importante mais c'est j'ai la Russie chez élargissement des critères extra-financiers n'est pas sans poser de difficultés. La première d'entre elles et la qualité de l'information donc financières dont disposent les investisseurs sur les structures dans lesquelles ils essaient ils investissent. Le règlement. Sf EDR. Rentrer en application en 2021 devrait permettre d'unifier cette documentation mais la marche à franchir pour les entreprises était grande et le calendrier très serré. La 2ème difficulté majeure réside dans une conception trop restrictive de la taxonomie européenne. Plusieurs secteurs font régulièrement savoir qu'ils éprouvent de grandes difficultés à trouver des financements. Je pense notamment à l'industrie de défense qui n'entrent pas dans les critères de la taxonomie européenne alors que le concours à l'indépendance. De notre pays, ainsi qu'à la défense de nos intérêts vitaux. Cette problématique que nous sommes ne concerne pas. Que des groupes intermédiaires depuis quelques années, certaines de nos plus grands groupes de défense je trouve en difficulté pour lever des financements. Par effet collatéral un risque de concentration de l'épargne ne donne des secteurs. Comme vers pourrait conduire à un sous-financement d'autres acteurs. Tout aussi importante pour l'économie française et européenne. Ma question est donc simple, Madame la Ministre dans quelle mesure le gouvernement peut-il favoriser l'accès des entreprises stratégiques à l'épargne privée, notamment dans le secteur de la défense et pour éviter que l'application des critères de la taxonomie conduisent à un sous-financement chronique de certains acteurs. Je vous remercie. Merci monsieur Maugars. Madame la Ministre pour la réponse. Merci. Madame la présidente, le sénateur Moga. Aborde dans la première partie de sa question. Le fameux. Si connu règlement essaie FDR mais ça fait plaisir d'en entendre parler parce que j'ai, il m'est arrivé d'être assez seul parfois pour en parler, y travailler donc. J'entends aussi la deuxième question mais je je veux déjà vous répondre sur la première, je suis restée FDR vous dire que. le cadre européen. Qui établit les les exigences spécifiques de reporting pour les acteurs financiers via ce règlement CFDA ou 10 clochard. S'inspire largement du 1er cadre français comme vous le savez. Établi par la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 au coeur de son article 173. La France est resté et a souhaité rester fer de lance sur le sujet et a adopté en 2021. L'article 29 de la loi énergie-climat et son décret d'application. Cadre réglementaire confirme la forte ambition en matière de finance durable et établi un un reporting plus ambitieux en particulier s'agissant de l'alignement des investissements sur les objectifs climatiques et de biodiversité, ainsi que j'aurai la gestion des risques. Le règlement est-ce FDR. Mériterait je vais parler au conditionnel parce que c'est une option que la commission est en train de regarder d'être. Renforcées et précisées. Il manque aujourd'hui. Un certain nombre de d'éléments et il est possible, on est en train de discuter avec la Commission européenne pour voir si nous pourrions reprendre ce règlement est-ce FDR et le préciser beaucoup plus fortement pour éviter. Que sous l'égide de produits financiers d'hiver on nous y mettent. D'autres actifs. Après vous mentionnez. Moi je vous réponds sur la partie vers des des des investissements et des investisseurs. Vous mentionnez un point très important. Qui est attention au risque d'éviction. Qui pourrait se mettre en, en, en place et Correa subir des industries stratégiques type défense. C'est une question, compte tenu du fait que j'ai déjà. Dépassé mon temps de 15 secondes à laquelle je propose de vous répondent par écrit, Monsieur le Sénateur Moga dans les jours qui viennent, je vous remercie. Merci madame la ministre, Monsieur. Vous ne souhaitez pas. Très bien. La parole est à monsieur Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains. Madame la présidente Madame la Ministre, mes chers collègues. Depuis plus de 20 ans, la France s'est engagée à développer ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises, en demandant aux entreprises de rendre des comptes sur autre chose que leurs performances financières. La loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a ainsi posé les premiers fondements du cadre législatif en matière de responsabilité sociétale des entreprises. Elle prévoit notamment que les entreprises cotées en Bourse indiquent dans leur rapport annuel. Une série d'informations relatives aux conséquences sociales et environnementales de leurs activités. Avec les lois Grenelle 1 et 2, le concept de RSE s'est démocratisé et s'est élargi à toutes les entreprises de plus de 500 salariés avec un bilan supérieur à 100 millions d'euros. Les exigences en matière de RSE n'ont eu de cesse de se renforcer, tant au plan national qu'européen. Afin d'accélérer le changement la commande publique a un rôle important à jouer. La loi de 2022 sur la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire impose désormais aux acheteurs publics un seuil minimal de 20% d'acquisition de produits issus du réemploi ou du reconditionnement. La commande publique a également été impactées par la loi dite climat et résilience de 2021. Ainsi, le plan national pour des achats durables. 2022 2025. A pour grand objectif d'accompagner les acheteurs publics dans la mise en oeuvre de cette loi. Les objectifs sont ambitieux, d'ici 2025 100 % des marchés publics devront intégrer des considérations environnementales et 30% devront comprendre des considérations sociales. Il ne fait aucun doute que la RSE n'a jamais été qu'un simple instrument de communication comme peuvent l'affirmer certains détracteurs mais elle constitue un levier de résilience qui permet à l'entreprise de se développer et de s'adapter à l'évolution de son environnement. Pour aborder notamment les nombreuses transition les critères ESG environnement social et gouvernance sont nécessaires. Pour autant, l'ARS ne doit pas être un synonyme d'un choc de complexité, comme les autres très bien le rapport d'information. C'est pourtant Suez craint de l'adoption par le Parlement européen le 10 novembre dernier de la directive sur la communication des données de durabilité 10 SRD élargissant l'obligation de diffusion d'informations, social et environnemental. Un grand nombre d'entreprises européennes. Qui n'était jusqu'alors pas concernés et notamment les PME. Ce sont donc environ 50.000 PME en plus des entreprises cotées en bourse qui devront se soumettre. À cette nouvelle directive légitimement il faut s'interroger sur la question de l'impact de cette décision sur les PME qui n'ont pas encore l'ingénierie nécessaires pour répondre à ces nouvelles obligations. L'ARS doit être intégrée au développement de l'entreprise mais ne doit pas la pénaliser imposer la RSE à marche forcée aux petites entreprises qui sont d'ailleurs souvent les plus vertueuses et contreproductif comme le stipule le rapport il est nécessaire de proportionner ces nouvelles exigences à la taille de l'entreprise. Enfin, je terminerai par rappeler combien la bataille des normes évoqués dans le rapport est crucial. Une domination des normes. Et d'une notation extra-financière américaine constituerait un véritable handicap pour les entreprises européennes. Comment imaginer que nos entreprises européennes soient jugés sur des critères non européens s'opposant parfois notre culture telles que des critères ethniques dans l'insertion professionnelle par exemple. Il faut donc aller vers des normes européennes. Qui opposeront qui imposeront Je terminale cette intervention, signalons que le modèle français est un modèle où la majorité des petites et moyennes entreprises repose sur un modèle de capitalisme familial. Ce que je vois d'ailleurs particulièrement dans mon beau département de la Mayenne.

veillons donc à continuer à les encourager dans ce sens et surtout ne pas les pénaliser sur un sujet sur lequel font déjà preuve de beaucoup de volontarisme, je vous remercie. Merci cher collègue. Madame la ministre vous avez la parole.

Et je pense qu'on est tous d'accord, je l'ai pas dit assez clairement, c'est vrai que la France est plutôt en avance en matière de responsabilité sociale des entreprises. Mais. Je crois que c'est une bonne raison pour contribuer à à. À la rationalisation. De la RSE au plan européen et donc l'idée c'est que. On a beaucoup de PME beaucoup de TI. Qui ont des pratiques en matière enfin qui ont des pratiques responsables tout simplement à l'endroit de leurs salariés à l'endroit de leur territoire à l'endroit de leurs fournisseurs à l'endroit de l'environnement. Mais c'est justement pour qu'on puisse mieux les valoriser et qu'on puisse mieux les comparer par rapport à d'autres PME européennes moins vertueuse que la France a intérêt assez SRD et j'assume. Totalement mon propos, je pense que c'est SRD est un outil. De compétitivité pour les entreprises européennes et pour nos PME aussi et j'ai parlé il y a quelques instants, en réponse à la sénatrice de proportionnalité de progressivité, donc ça n'est ni le même calendrier, ni les mêmes indicateurs en terme de profondeur et d'ampleur de travail. Qui seront demandés à nos PME. Et je rappelle que le Champ de la directive ne concerne que les PME cotées et qu'il peut y avoir des incidences. Dans le cas de la chaîne de sous-traitance mais que les PME cotées seront les seuls concernés. Je vous dis ça parce que. Ça n'a pas été votre cas. Monsieur le sénateur, mais il arrive parfois qu'on on se fasse peur. Les PME non cotées françaises. Ne seront pas contraintes par les 80 indicateurs macro-sectorielles portées dans CSR des on a assez de raisons de d'être angoissé. Pour ne pas s'angoisser en plus pour ça. Et elles ont. Plutôt de l'avance et j'aurai l'occasion d'en dire un mot dans la conclusion dans quelques minutes. Elles sont plutôt à Londres. Vous l'avez rappelé, et pas que les PME familiale, on a un don, un code du travail qui est quand même assez exigeants dans notre pays on n'a. Pas vraiment de retard en matière de considérations environnementales et on est plutôt sur la balle sur le sujet de la gouvernance. Donc on a plutôt notre épingle à tirer nos PME aussi. De cette législation. Je, j'ai donc. Pas d'autres les éléments à vous apporter, si ce n'est que cette considération de la taille de l'entreprise sur Madame les la progressivité. Et la proportionnalité sont acquises. C'est des choses qu'on a gagné au vote de la directive en le 24 février dernier. Donc à nous de le mettre en oeuvre, on a cinq ans pour le mettre en oeuvre sur nos PME cotées et je pense qu'on est tout à fait capable de le faire, à voir comment on accompagne au mieux ce sera l'objet de ma prise de parole dans la conclusion. Merci, madame la Ministre bé écoutez. Je vous propose d'enchaîner tout de suite sur la conclusion

Madame messieurs les les sénateurs. Pour la réalisation de ce rapport. Mais aussi oui. Monsieur le président de la délégation aux entreprises, Monsieur le Sénateur. Babary. Je veux vraiment d'abord vous remercier pour la qualité de ce rapport. Pour votre. Votre. Détermination à l'endroit de la RSE, année après année. Et me réjouir aussi. Du fait que malgré des divergences politiques et ça enrichit le débat on partage quand même les même constats. Et nous partageons aussi je crois les mêmes préoccupations. Et pour la plupart d'entre vous. Aussi bien souvent les mêmes moyens, les mêmes objectifs. Nous sommes d'accord je crois sur l'importance pour ne pas dire sur l'urgence de la transition écologique sociale mais aussi de gouvernance de nos entreprises. Une fois qu'on a dit ça je vous le disais au démarrage il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que nous sommes en train de construire des outils. Dont on ne sait pas encore, au moment où on se parle s'ils seront parfaitement opérant face aux défis immenses que pose l'adaptation de nos sociétés. Nos économies à la nouvelle donne climatique et mon ange. À l'époque en tant que secrétaire d'État à l'économie responsable c'était justement de faire en sorte que les entreprises puissent. Proposer. Puissent. Être force de proposition et mon ange désormais en tant que ministre déléguée en charge des PME, c'est de faire en sorte que toutes les entreprises puissent adopter. Ces nouvelles règles du. Je reprends à mon compte l'expression qui a été employé par plusieurs d'entre vous. La réglementation extra-financière telle que se présente aujourd'hui à des non-initiés. Ce qui est, ne nous voilons pas la face. La situation d'une immense majorité de nos entreprises, de nos PME notamment représente et je reprends l'expression, un choc de complexité cette complexité. C'est une évidence aujourd'hui. Mais tout l'enjeu, c'est que ce ne soit pas une réalité demain cette complexité. Vous l'avez dit, les PME ne sont pas directement concernés. Je vous l'ai redit à quelques instants dans la plupart des réglementations actuellement en construction. Et si les PME ne sont pas directement concernés. Il faut admettre et je crois qu'on est plusieurs à l'admettent qu'elles vont l'être indirectement. Structurellement, parce que la transition écologique, suppose un changement de modèle, et donc de toutes les entreprises, pas uniquement les plus grandes socialement parce que la demande des consommateurs pour des biens, des services plus durable et concerne mais aussi parce que pour faire tourner nos belles entreprises il faut des salariés et vous l'avez mentionné notamment madame la sénatrice y a quelques instants, les jeunes salariés. Ne n'arbitre par qu'à l'aune de la performance financière. Les entreprises dans lesquelles ils ont envie d'aller. Travailler il la RSE est un enjeu d'attractivité majeure dans la bataille des compétences que nos PME doivent continuer à gagner et je suis parfois inquiète ça n'a pas été le cas ce soir et je vous en remercie. Quand j'entends des discours un peu radicaux de surtout pas nos PME. Et nous aurons des débats dans disons ici même où on se dira mais. Quelle mouche vous avez piqué pour laisser les PME à côté de cette révolution environnementale, sociale et de gouvernance parce que le cas échéant nous arriverions dans 10 15 ans à des entreprises à 2 vitesses à 2 visages et donc des entreprises qui pour certaines ayant une politique de RSE réelle et tangible attirer les talents et à côté des PME dont nous savons pertinemment qu'elle manque déjà de compétences qui se retrouveraient sur le le côté du chemin. Moi c'est un, un sujet en tant que ministre délégué aux PME qui m'interpelle tout particulièrement je sais que c'est plus compliqué pour nos PME. Mais je sais aussi que ne pas le faire serait irresponsable ne pas embarquer, nos PME dans. Le le la révolution de l'extra financiers et de la responsabilité sociale des entreprises seraient quelque part condamné ou insulter une partie de leur avenir. Mais aussi au plan juridique. Enfin. On se les dit rapidement parce que beaucoup de TPE de PME ont des donneurs d'ordres qui vont réclamer de plus en plus d'informations au plan environnemental, social. Dans le cadre de la chaîne de valeur. Alors je voulais vous dire que. J'ai demandé à la direction générale des entreprises de travailler à l'amélioration. De la plateforme impact Point gouv Point FR que je chéris parce qu'on peut chérir des plateformes et je chéris cette plateforme impact Point gouv Point FR que j'ai lancé il y a un peu plus d'un an. Et d'ailleurs on m'avait dit à l'époque. Au-delà du fait. Ça ne marcherait jamais qu'il n'y aurait pas de PME. Prenez le temps d'aller voir je vous en supplie, Mesdames, messieurs les sénateurs, la majorité sont plutôt des PME sur cette plateforme des PME qui donne des informations celles qu'elles peuvent sur leur bilan carbone sur leur bilan social et qui aujourd'hui jouent le jeu de la transparence en matière de responsabilité sociale des entreprises, j'ai proposé la DGE d'en faire l'outil public de référence. Pour permettre aux entreprises de se conformer à la réglementation en simplifiant leur parcours mais aussi. En les accompagnant avec les administrations notamment pour nos PME. Cette plateforme, elle va évoluer et elle va devenir une plateforme d'accompagnement dans le cas de tous les référentiels aujourd'hui devenu qui vont devenir obligatoires pour nos entreprises de taille intermédiaire mais aussi pour nos PME. Et c'est donc. Une nouvelle version d'un. Point gouv point FR qui va se déployer dans les prochains mois. Ça n'est pas parce que j'ai changé de poste que je ne suis pas attentivement cette plateforme et elle va continuer à évoluer avec la DGE pour mieux accompagner nos entreprises notamment nos PME qu'elle soit d'ailleurs côté ou non. J'aurai à coeur d'ailleurs de vous en reparler. Si ça vous intéresse dans les prochains mois parce que c'est une évolution qu'on met en oeuvre avec la DGE. Je vous remercie et pardon de mai 51 secondes de retard sur le temps. Merci madame la ministre. Et pour conclure le débat. La parole est à monsieur Serge Babary, président de la délégation sénatoriale aux entreprises.

Madame la présidente, madame la Ministre. La qualité. Des échanges et des interventions justifie. Le fait que nous ayons portées. Au débat. Les conclusions de notre rapport. Il est vrai que. Nous nous intéressons. Depuis quelque temps déjà à la RSE. Ainsi que l'ont rappelé nos nos rapporteurs à l'introduction, la délégation aux entreprises s'est intéressé à deux reprises dernièrement en juin 2020 et en octobre dernier. À la responsabilité sociétale des entreprises. Je rappelle que dès 1972. Antoine Riboud, PDG de Danone. Expliquer aux Assises nationales du CNPF à l'époque que la responsabilité de l'entreprise ne s'arrête au seuil des usines ou des bureaux. Son action se fait sentir dans la collectivité toute entière et influe sur la qualité de la vie de chaque citoyen. 30 ans après, la même définition était reprise par la Commission européenne dans son livre Vert de juillet 2001. La France s'est voulu et a été pionnière en la matière. En portant l'Union européenne vers une nouvelle définition de l'entreprise. Ce mouvement s'est cependant traduit parallèlement par une accumulation de normes volontaires et légale européennes et nationales visant principalement les grandes entreprises d'abord côté mais ensuite par lui seulement les ETI et les PME. Notre collègue Martine Berthet. On a décrit pertinemment le processus. A les émetteurs de normes environnementales, sociales et de gouvernance ESG résonne verticalement et produisant silos tandis que le chef d'entreprise et souvent bien seul, surtout dans une PME avec d'autres préoccupations et priorités. Qui a chiffré le coup organisationnels humains et financiers de ces normes qui individuellement sont toutes justifiées mais qui alignait cumuler sédimentaires sont en capacité d'affaiblir la compétitivité de nos entreprises, surtout si leurs concurrents non-européens s'en exonère. Certes la RSE, est un atout. Elle devient un critère désormais déterminant des investisseurs, même si la finance verte restent encore bien grise comme l'a souligné, notre collègue Florence Patrice content mais la nécessité de simplifier et d'harmoniser et d'adapter, notamment pour les PME, évoqué dans le 1er rapport de la délégation des 2020 reste plus que jamais d'actualité. Plus généralement, la simplification de notre appareil administratif et de nos normes économiques ou financières. Doit redevenir une politique publique. C'est la raison pour laquelle la délégation lance un nouveau cycle d'auditions sur ce sujet. Les entreprises attendent toujours un vrai choc de simplification. Je sais que vous y êtes extrêmement sensible. Avec la loi pacte les entreprises se sont vu proposer une sorte de statut RSE pour transformer leur nature juridique afin de prendre en considération les impacts tant positifs que négatifs sur leur partie prenante. Il faut les protéger dans cette démarche. C'est pourquoi nous avons proposé dans le rapport d'octobre 2022. Qu'un investisseur puisse être obligé de préciser ses intentions lorsqu'il conteste la démarche RSE d'une société. Afin de permettre à cette dernière d'accélérer l'alignement de sa stratégie sur les objectifs ESG qu'elle se propose d'atteindre. Je me réjouis de constater que le Club des juristes a rejoint les conclusions de la délégation d'entreprises dans la mise à jour de décembre. Décembre 2022, de son rapport de 2009 sur l'activisme actionnarial. Il suggère que l'AMF propose une recommandation visant à ce que tout investisseur prenant des positions publiquement en vue d'influencer la stratégie, la situation financière ou la gouvernance d'un émetteur, déclare ce niveau de participation à l'émetteur et plus généralement au public au-delà des obligations déclaratives résultant d'un franchissement de seuil. Nous avons tous en mémoire l'affaire Danone. Elle a été cité engagés dans une démarche RSE qui a déplu à des fonds activiste craignant un moindre profit. Je rejoins également notre collègue Jacques Launay. Quant à la nécessité d'une harmonisation mondiale des normes ESG sans sacrifier la double matérialité qui est une véritable valeur ajoutée européenne dans ce but, ce dossier doit être porté au plus haut niveau de l'État et bénéficier d'un suivi attentif du Conseil européen. La maîtrise des émissions carbone et la comptabilité extra-financière reste à construire. L'Union européenne le peut se défausser sur des acteurs privés a fortiori américain pour les définir. Il en va de la reconquête de notre souveraineté économique. Ce sont à ces conditions simplification consolidation unification. Que l'ambition de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises doit pouvoir devenir un atout pour chaque entreprise française ou européenne, quelle que soit sa taille, je vous remercie. je vous remercie. Mes chers collègues, je vais lever la séance. Prochaine séance mercredi 11 janvier à 15h pour les questions d'actualité au gouvernement. La séance est levée.